La séance est reprise. L’ordre du jour appelle la nomination des membres des sept commissions permanentes et de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l’évaluation interne. Conformément aux articles 8 et 103 du règlement, la liste des candidats remise par les présidents des groupes et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe a été publiée. Je rappelle que, en application de ce même article 8, la répartition des sièges au sein des commissions permanentes se fait dans le respect de la proportionnelle au plus fort reste.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance fixée à demain, jeudi 5 octobre, à quatorze heures trente : Annonce de la publication des listes des candidats à la commission des affaires européennes et à la commission spéciale sur le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, et de leur ratification, sauf opposition dans le délai d’une heure. Nous resterons